La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 23 janvier 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le

je tiens, en votre nom, à associer notre Haute Assemblée aux commémorations marquant le 75 anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. ans après, nous avons le devoir de rappeler la monstruosité de ces crimes et de maintenir le souvenir des victimes : 6 millions de morts sur notre continent 76 000 Juifs déportés de France, dont les noms sont inscrits, au Mémorial de la Shoah, sur le Mur des noms. Au-delà de la commémoration, il nous revient aujourd'hui de continuer à faire vivre la mémoire de l'Holocauste pour ne jamais oublier. Face à la montée de l'antisémitisme à travers le monde et à l'augmentation du nombre d'actes racistes et xénophobes dans notre pays, il nous faut plus que jamais nous souvenir et demeurer vigilants. Restons unis et intransigeants face à l'antisémitisme, au racisme, à la xénophobie et à l'intolérance. La conférence des La conférence des présidents, qui vient de se réunir, a décidé de s'opposer à l'engagement de la procédure accélérée sur le projet de loi organique relatif au système universel de retraite et sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Cette décision sera notifiée à M. le président de l'Assemblée nationale. Acte est donné de cette communication. communication. La conférence des présidents a pris acte, en application de l'article 6 du règlement, de la demande du groupe CRCE de création d'une mission d'information sur le thème Quel rôle, quelle place, quelles compétences des départements dans les régions fusionnées, aujourd'hui et demain ? » La désignation des membres de cette mission en séance publique interviendra le mercredi 19 février, à seize J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique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

spéciale, d'une demande de priorité sur l'article 17, afin qu'il soit examiné avant l'article 14. Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Cohen, sur l'article. Nous voterons cet article sur le don du sang et je voudrais en profiter pour dire quelques mots sur le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), créé en réponse à l'affaire du sang contaminé. Le LFB, qui conçoit et fabrique des médicaments à partir de plasma, est détenu pour l'instant à 100 % par l'État. Malheureusement, il semblerait que des menaces pèsent sur cette maîtrise publique puisque des investisseurs privés pourraient entrer dans le capital de cette entreprise. Je ne méconnais pas les difficultés financières du LFB et son plan stratégique de transformation, mais, madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer et nous indiquer si la participation de l'État va continuer à être à hauteur de 100 % ? Je suis déjà intervenue, à plusieurs reprises, vous le savez bien, pour défendre cette participation essentielle de l'État. Les raisons en sont simples : si l'État ne détient pas cette majorité, c'est la porte ouverte à la marchandisation du don du sang, remettant en cause les principes éthiques de gratuité de ce don,

Donner son corps à la science est un geste tout à fait exceptionnel, mais, néanmoins, fondamental pour la recherche et la formation, notamment dans le domaine médical. Les modalités du don sont bien établies depuis une loi de 1887, qui dispose que le don est issu de dispositions testamentaires. Pour autant, si la manière dont on fait le don de son corps à la science est bien encadrée, ce qu'il en advient ensuite ne l'est pas suffisamment. L'actualité récente l'a mis en évidence. Une mission toujours en cours,

En 2017, 27 centres de dons ont reçu les corps de 3 400 donateurs. Au-delà des chiffres, chacun comprend naturellement la nécessité, ne serait-ce que sur le plan éthique,

et de renvoyer à un décret en Conseil d'État des dispositions réglementaires propres à l'organisation de ces centres. Cet amendement nous permettra ainsi de garantir le plus haut degré d'exigence éthique que nous devons aux donneurs, à leurs familles, aux chercheurs et aux étudiants. Je vous invite donc à le voter. Quel est

Cela dit, il apparaît effectivement souhaitable d'offrir un cadre législatif au don de corps à des fins d'enseignement médical ou de recherche, qui est, pour l'heure, simplement régi par un article de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Avec l'article 3, nous avons autorisé la levée de l'anonymat pour les enfants nés de dons de gamètes. Cette évolution pose la question de la levée de l'anonymat pour les enfants nés d'un accouchement sous le secret. Certes, les situations ne sont pas comparables et mon objectif, au travers de cet amendement, n'est pas de nier cette différence. Néanmoins, en levant l'anonymat pour les enfants nés de dons de gamètes, on suscite une interrogation, voire une incompréhension, pour ceux qui sont légitimement se demander : « Pourquoi pas nous ? » D'autant que les arguments qui ont prévalu pour la levée de l'anonymat pour les enfants nés de dons de gamètes peuvent également être mis en avant pour ceux qui sont L'intérêt supérieur de l'enfant dans sa recherche d'identité se double d'une recherche de sens, pour comprendre ce qu'il a vécu de sa conception à son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et dont nul ne peut ignorer les conséquences sur le reste de sa vie. Le développement des grandes bases de données génétiques, comme l'expliquait la semaine dernière Gérard Longuet, fait qu'on peut aujourd'hui, par ces voies-là, découvrir son identité. J'ajoute un argument en faveur de cet amendement à l'article 9 : l'argument de santé publique. Cet article permet en effet aux enfants nés de dons de gamètes de prévenir les donneurs d'une maladie génétique pouvant être responsable d'une infection grave. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les mères qui ont eu recours à un accouchement sous le secret et aux enfants qui en sont nés ?

dans le secret. C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur cet amendement, qui, par ailleurs, tend aussi à supprimer le caractère automatique personnelles) pour la transmission d'une information d'ordre médical entre une personne née dans le secret et l'un des parents de naissance en cas de détection d'une anomalie génétique potentiellement grave. Le cas échéant,

au personnel soignant de l'équipe gynécologique des informations sur leur situation, toujours singulière, toujours douloureuse. Il ne faudrait pas, au travers de cet amendement à faciliter les recherches génétiques de la mère vers l'enfant, de revenir sur cet équilibre entre le droit des femmes de pouvoir accoucher de manière anonyme et le droit de l'enfant de pouvoir

des caractéristiques génétiques. Nous visons ici davantage les tests dits « récréatifs », qui se multiplient notamment les réseaux sociaux, pour soi-disant connaître la diversité de ses origines. Nous avons, bien sûr, entendu les arguments développés par le rapporteur et ceux qu'a exposés Mme la ministre, notamment en séance à l'Assemblée nationale. Mais il nous semble que, au contraire, ces précisions ne sont pas satisfaites par le code en Comme vous l'avez expliqué en octobre dernier, madame la ministre, un annonceur étranger a diffusé, à l'été 2018, sur plusieurs chaînes de télévision, une publicité pour les tests ADN, et vous aviez indiqué que le Conseil par la suite adressé aux chaînes concernées une mise en garde. La publicité avait alors été retirée. Malheureusement, les démarchages fleurissent toujours, particulièrement sur les réseaux sociaux, en toute impunité. Nombreuses sont nos concitoyennes et nombreux sont moyennant quelques euros, qui envoient des données personnelles, qui sont stockées dans un pays étranger- avec quelle finalité ? On peut avoir bien des craintes -et qui reçoivent ensuite une fiche qui établit la composition, notamment géographique, de leur profil. Au moment où l'on parle d'éthique, il nous semble, au groupe CRCE, que cela pose question ! Je crois qu'il est de notre responsabilité, d'une part, d'informer sur les dangers et dérives éventuelles, d'autre part, et surtout, de faire en sorte que ces publicités soient interdites et que les entreprises concernées soient sanctionnées

de l'interdiction de la commercialisation de tests génétiques. Nous assistons aujourd'hui à une recrudescence des entreprises privées étrangères proposant des tests génétiques en libre accès sur internet malgré leur interdiction actuelle en France, là encore sans que nous soyons en mesure de connaître le sort de ces données

Je souhaite exposer les raisons qui amènent le Gouvernement à être profondément défavorable à cette possibilité. Le législateur a circonscrit, dès les premières lois de bioéthique de 1994, le recours aux examens génétiques. Ainsi, les finalités de ces examens sont limitées ces tests peuvent être entrepris uniquement à des fins médicales ou de recherches scientifiques ainsi qu'à des fins judiciaires. Des garanties spécifiques entourent la réalisation de ces examens, quelles qu'en soient les finalités. le cadre est médical, le parcours de soins est très encadré et la discussion entre le médecin et le patient qui réalise le test est au coeur du processus. En recherche, les contraintes spécifiques pèsent sur les chercheurs, comme cela apparaît à l'article 18 de ce projet de loi. Lorsque ces tests sont effectués à des fins judiciaires, seul un juge peut en ordonner la réalisation dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire. Par ailleurs, toute discrimination sur des caractéristiques génétiques est bien entendu interdite, notamment dans le cadre des relations de travail. Les banques et les assurances ne peuvent pas prendre en compte ces caractéristiques, même si elles leur sont volontairement transmises par la personne concernée. Je sais que ces tests génétiques, généalogiques, connaissent un fort développement à l'étranger et que certains de nos concitoyens y ont recours, malgré leur interdiction en France. Ces tests exposent à une multitude de risques peu connus, qui constituent toutefois une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs. Les premiers risques qui peuvent être cités sont liés à l'incertitude sur la précision et la fiabilité des résultats obtenus. La qualité des résultats dépend des bases de données de référence utilisées pour comparer l'ADN avec un ADN de référence. Cela dépend notamment des tailles des échantillons dont disposent ces industriels, des types de population dont ils disposent dans leur base de données, des critères mobilisés pour créer des catégories, qualifier et délimiter des groupes de comparaison. Cela dépend aussi évidemment des algorithmes qu'ils ont mis au point. Cela explique les différences de résultats que l'on obtient en fonction de la marque du test Même les meilleures bases de données actuelles ne représentent qu'un échantillonnage très médiocre de la diversité génétique humaine mondiale. Ce manque de fiabilité transparaît dans les divergences de résultats obtenus pour un même ADN qui est envoyé à différents laboratoires. Par ailleurs, les résultats obtenus sont potentiellement trompeurs, à tout le moins purement indicatifs. En effet, l'utilisation de populations contemporaines et non ancestrales pour la comparaison avec les ADN individuels testés ne fait qu'ajouter à la complexité des résultats et à leur interprétation. Ces tests sont abusivement appelés tests d'origine ou d'ancestralité, mais ne révèlent pas d'où vient notre ADN dans le passé. Ils révèlent plutôt dans quelle mesure il ressemble à des ADN présents aujourd'hui sur la planète.

Ces tests sont également parfois utilisés à partir des données recueillies et exploitées à des fins commerciales. Nous ne sommes donc pas sûrs du respect de la protection de la vie privée, pas plus que de la confidentialité des données et il y a un manque de clarté sur les conditions générales de vente.

d'autres usagers qui leur sont génétiquement similaires ou de préciser, pour chacun, leur degré de parentalité. Si cette recherche est utilisée par les personnes conçues à partir d'un don de gamètes ou de personnes adoptées nées sous X souhaitant, à partir d'une enquête généalogique et de déductions, retrouver leurs origines biologiques, ce service conduit parfois à des révélations inattendues au sein des familles, d'autant que les autres membres de la famille qui peuvent partager ce patrimoine génétique ne sont pas informés de la réalisation de ces tests et n'y ont donc pas consenti. En outre, ces tests peuvent être volontairement détournés pour confirmer ou infirmer une paternité ou des liens de parenté. Aux États-Unis, le Pentagone a également pris position sur ces tests, les militaires ayant fait l'objet de publicité de la part des sociétés qui les commercialisent. Une note visant à mettre en garde les soldats américains contre leur utilisation leur a été adressée par le secrétaire adjoint de la défense pour le renseignement. Elle mérite que l'on s'y attarde. Cette note prévient que les tests ADN commerciaux, particulièrement non régulés, sont de nature à révéler des informations personnelles et génétiques, et pourraient avoir des conséquences imprévues pour les forces armées et leurs missions, ainsi que sur la carrière des militaires américains. Elle précise également que l'exposition d'informations génétiques sensibles à des tiers pose des risques personnels et opérationnels. La crainte des responsables du Pentagone est de voir tomber les données génétiques de ces soldats entre de mauvaises mains. Cette note explique encore que la communauté scientifique est de plus en plus préoccupée par le fait que des tiers exploitent l'utilisation des données génétiques à des fins discutables, y compris la surveillance de masse et la possibilité de suivre les individus sans leur autorisation ou sans qu'ils en aient connaissance. Par ailleurs, ces tests sont susceptibles de déceler de manière involontaire des marqueurs de certaines maladies et affections génétiques qui pourraient finir par affecter la carrière d'un militaire, comme celle de chacun d'entre nous, a commenté un porte-parole du Pentagone. vous le comprenez : le risque est réel. Il est grave. Il constitue une véritable menace pour nos sociétés. L'ADN est une donnée fort utile pour qui cherche à trier, sélectionner, discriminer et assigner à des individus une identité figée sur la base d'informations biologiques pouvant être présentées comme scientifiques. Si la lecture de la séquence d'un génome humain ne pose aucune difficulté- elle est même clairement démocratisée, si je puis dire -, son interprétation reste très complexe et dépend notamment des bases de données auxquelles on compare le génome ou les parties du génome que l'on examine. Elle doit être justifiée par des objectifs légitimes, notamment médicaux, et ne peut l'être uniquement par un pseudo-intérêt récréatif, qui peut entraîner des conséquences néfastes pour l'intéressé comme pour sa famille. Il nous semble que ces tests n'ont de récréatif que le nom. Il n'y a pas de situation simple avec les tests génétiques. C'est pourquoi leur réalisation est très encadrée et très accompagnée en France. À cet égard, il faut rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son étude « bioéthique » de 2018, que l'interdit visant des assurances « serait plus difficile à préserver dès lors que l'accès à l'information serait libéralisé et le séquençage banalisé Nous devons nous positionner de façon rationnelle et raisonnable pour la responsabilisation des professionnels intervenant dans ce secteur, comme des consommateurs parfois attirés par ces nouveaux produits, en prenant en compte notre modèle bioéthique à la française, qui protège avant tout les droits et la liberté des individus.

C'est en garantissant ces limites aujourd'hui que nous pourrons ouvrir demain des développements, notamment issus d'une recherche bien encadrée, qui seront véritablement source de progrès médical et scientifique pour nos concitoyens. Mesdames, messieurs les sénateurs, pour toutes

Le débat n'est pas de savoir s'il faut qu'ils existent ou si l'on doit favoriser leur existence : ils existent. Aujourd'hui, je fais référence à un débat précédent, l'interdiction des tests génétiques en accès libre sur internet est

d'informations médicales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les données du million de Français qui ont eu recours à ces tests sans aucun encadrement sont envoyées dans la nature sans aucun contrôle.

après avoir réalisé un test ADN généalogique. La journaliste de France 2 faisait d'ailleurs remarquer que cette pratique était interdite en France, mais la société installée aux États-Unis échappe

à l'étranger- aux États-Unis, en Israël ... -des tests de cette nature par le biais de sociétés qui, de ce fait, détiennent des informations et qui les utilisent selon leur législation nationale, et pas selon la nôtre.

vraiment favorable à ce que l'on s'en tienne à l'encadrement actuel. Ces examens ne sont justifiés qu'à des fins médicales et, évidemment, judiciaires, vous l'avez rappelé,

Ce dispositif sera parfaitement inefficace. Pourquoi ? Parce que, chaque année, environ un millier d'enfants naissent avec une maladie génétique grave et incurable. Or, neuf fois sur dix, il n'y a pas d'antécédent dans la famille. J'ajoute que le dépistage préconceptionnel ne peut en aucun cas prévenir des maladies liées à des mutations, c'est-à-dire qui surviennent par hasard au moment de la conception, sans être présentes dans le génome des parents.

des Français qui font appel à ces tests. C'est dans cet esprit que nous avions rédigé cet amendement et que le rapporteur a avancé ses explications. Mes chers collègues, il ne s'agit pas ici d'autoriser quelque chose qui se fait ailleurs : il s'agit de permettre que les Français qui sollicitent ces tests ailleurs

À quoi sert-il de poser des interdits si nous n'arrivons pas à les faire respecter ? Il vaut peut-être mieux, dans ces cas-là, protéger nos concitoyens. Enfin, madame la ministre, vous m'avez rassuré sur un autre sujet. Vous avez évoqué l'avis du Conseil d'État. Votre intérêt pour le Conseil d'État me fait penser que vous allez changer d'avis sur les retraites

savons très bien que cela ne s'arrêtera pas, que nous n'aurons pas les moyens de l'arrêter et que ces tests vont se développer. En pensant faire du mieux-disant éthique, on livre nos compatriotes à du moins-disant, c'est-à-dire aux règles qui sont appliquées ailleurs, où il n'y a pas

explication de vote. On parle ici des tests ADN généalogiques. Or j'entends que ce serait une activité récréative.

sont à la recherche de leurs origines et qui, déjà depuis des années, comme cela se fait dans le monde entier, recourent à des prestataires qui se trouvent à l'étranger, continueront à le faire, et ce pour une raison très simple simple : les recherches généalogiques sont beaucoup plus efficaces lorsque l'on s'adresse à une banque de données qui regroupe des millions de données plutôt qu'à une société débutante.

loin de devenir les auxiliaires d'entreprises qui voudraient prendre position sur un marché prometteur, défendre

Que de précautions avons-nous voulu prendre pour protéger nos données, qui étaient essentiellement des données matérielles, mais qui concernaient notre vie privée ! ce sont plus que des données matérielles. Ce ne sont pas des questions de patrimoine ou d'argent. Ce sont des questions qui touchent à nos origines, qui sont véritablement au coeur de notre vie personnelle.

à consulter des sites étrangers pour avoir l'assurance d'accéder à des bases de données beaucoup plus volumineuses. La prudence, c'est de dire à nos concitoyens : « Chers concitoyens, ne faites pas des tests génétiques au prétexte que vous êtes curieux de votre histoire, car vos données génétiques vont se balader dans le monde entier et vous ne savez pas ce que l'on en fera.

à des changements de comportement et de législation, et que chaque Français pourra accéder à des données peu fiables, potentiellement médicales.

mais peut-être aussi une maladie potentiellement grave et mortelle à l'âge de 5 ans, ou une maladie grave, pas mortelle, mais responsable d'un handicap à vie, ou une maladie mortelle à l'âge de 30 ans ou un Alzheimer à 40 ans. Qui fixera la limite ?

Je suis intimement persuadée qu'il pourrait changer les comportements des jeunes couples, avant même le mariage. Je pense que tout le monde se sentira dans l'obligation un jour de faire des tests pour s'assurer que son enfant ne sera pas porteur du gène de telle ou telle pathologie.

bien. Cela donne l'image d'une société où le génome détermine tout, où l'humain contrôle sa descendance. C'est le mythe de générations futures indemnes.

actuelle, qui prévoit que tout test génétique doit considérer un risque unique, dans une famille unique, dans le cadre d'un parcours de soins, sur prescription médicale.

les effets d'analyses génétiques sur les générations ultérieures. Il me semble que l'article adopté en commission spéciale donne une vision de la société

Il nous a semblé que la dérive eugénique n'était pas constituée puisqu'il ne s'agit pas de sélection d'embryons. En effet, l'examen génétique envisagé n'intervient pas dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Aucun embryon n'a donc été conçu au stade de cet examen, que ce soit naturellement ou par AMP. Il s'agit en réalité pour une personne de déterminer si elle est porteuse ou non d'une mutation génétique grave et d'évaluer le risque que cette mutation puisse donner lieu à une pathologie, ou que cette mutation puisse se transmettre aux enfants. Lors de leur audition par la commission spéciale, les professionnels ont insisté sur le fait que certaines pathologies graves, comme la mucoviscidose ou l'amyotrophie spinale infantile, infantile, survenaient souvent chez un enfant sans que les parents sachent qu'ils étaient tous les deux porteurs de cette mutation, faute d'antécédent familial.

a indiqué : « Si nous pouvions, comme dans de nombreux pays, proposer aux jeunes couples de rechercher les principales anomalies génétiques pour leur éviter l'interruption de grossesse, soit en proposant un diagnostic préimplantatoire soit pour envisager une grossesse spontanée,

plus de connaissances, mais je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre ce que la recherche veut, ce qu'elle permet, et ce qu'il y a de mieux pour la société et les êtres humains dans leur individualité.

l'eugénisme sélectionne à partir de caractéristiques ; la médecine, elle, donne les moyens d'éviter des maladies et des pathologies. Certes, la frontière n'est pas évidente, j'en donne acte à chacun dans cette assemblée. Et il est complexe pour le législateur de fixer la frontière. Cela

10 : « [ ...] Après consultation de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des sociétés savantes en génétique médicale, les anomalies génétiques susceptibles d'être recherchées dans le cadre de cet examen peuvent être limitées à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.

peut être faite « par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique sans qu'il soit nécessaire pour la personne qui en fait la demande de présenter les symptômes d'une maladie à caractère génétique ou de faire état d'antécédents familiaux d'une telle maladie ». Il est ensuite précisé

pouvant être responsables d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins ». Ainsi, on ne recherche plus d'antécédents familiaux, et un médecin décide de rechercher quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il prescrit- on ne sait pas en vertu de quoi

ainsi, après consultation « de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des sociétés savantes », il est prévu « une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche ». Mais, mes chers collègues,

à tester leurs génomes avant de faire un enfant et à vérifier si dix gènes ou vingt gènes sont présents chez le père ou la mère. Dans ce cas, on leur donne un conseil génétique, on trie les embryons et on leur garantit un enfant sans

Je ne pense pas que ce soit aux experts aujourd'hui de décider quel type de société nous souhaitons et de définir une liste de ce qui est acceptable ou pas.

par rapport à ce qui se passerait.

Cela n'a rien à voir avec la trisomie 21, qui n'est pas une maladie génétique ; c'est une anomalie acquise. Elle est dépistée uniquement chez les femmes déjà porteuses de l'enfant. Je

abyssales. Je ne sais pas pourquoi je laisserais à des généticiens, à des obstétriciens ou à des pédiatres le choix de décider que la souffrance physique, la souffrance psychique, la mort à 5 ans ou la mort à l'âge de 10 ans

Je considère qu'on ouvre la porte à un champ des possibles effrayant : on commence par trois maladies graves mortelles à l'âge de 1 an et, dans dix ou vingt ans, on refusera des maladies trop coûteuses à l'âge de 30 ans.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

à se tourner vers d'autres solutions conçues hors d'Europe, dont nous ne pourrions garantir le caractère éthique. L'article 11 introduit donc trois nouvelles normes nécessaires un devoir d'information du patient sur le recours à l'intelligence artificielle dans sa prise en charge ; un nouveau principe, fondamental, de garantie humaine de l'intelligence artificielle, permettant d'assurer que l'algorithme et son évolution resteront sous la supervision de professionnels de santé ; enfin, une obligation de traçabilité tout au long du processus de médecine algorithmique. Il me semble que ces normes apportent des garanties suffisantes. Depuis sa reconnaissance par le CCNE, le principe de garantie humaine de l'intelligence artificielle en santé a été repris en Europe,

Le moment est à la préparation active de sa mise en oeuvre par un effort résolu de formation des professionnels médicaux et paramédicaux aux potentialités nouvelles, mais aussi aux risques éthiques associés à la diffusion de l'IA en santé. Il ne faut plus différer cette nécessaire préparation collective !

En la matière, le rapporteur en charge de cette problématique a fait un travail qui, selon nous, va dans le sens du respect de nos principes éthiques, notamment avec la consécration du principe d'une garantie humaine dans l'interprétation des résultats en cas d'utilisation d'un algorithme. En ce sens, certaines recommandations de la CNIL, du CCNE et du Défenseur des droits ont été prises en compte. D'autres, en revanche, ont été laissées de côté. Nous souhaitons les intégrer au texte de la commission

algorithmique des données sanitaires, dont il nous semble important de ne pas faire l'économie.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

J'ai demandé que soit examiné en priorité l'article 17, car il aborde la question fondamentale des interdits. La définition de ces derniers, s'agissant notamment des embryons chimériques, aura nécessairement un impact sur l'encadrement qui nous semble le plus opportun pour les recherches sur l'embryon et les cellules souches, traitées aux articles 14 et 15. Avant d'aborder l'article Avant d'aborder l'article 17, permettez-moi de clarifier les termes du débat autour des embryons chimériques, en rappelant ce qui est aujourd'hui interdit et ce qui ne l'est pas. L'interdiction des embryons chimériques figure dans le code de la santé publique. Deux types de chimères sont aujourd'hui interdits : d'une part, la modification d'embryons humains par l'insertion de cellules animales ; d'autre part, la modification d'embryons animaux par l'insertion de cellules souches embryonnaires humaines. En revanche, rien ne régit les chimères à partir de cellules souches pluripotentes induites humaines, les fameuses cellules iPS. Ce silence de la loi permet actuellement d'expérimenter l'insertion dans un embryon animal de cellules iPS humaines : ce sont les seuls embryons chimériques possibles en France, expérimentés par des équipes françaises à partir d'embryons de lapins et de macaques. Que propose le projet de loi du Gouvernement ? Il va résolument plus loin que ce qui est possible aujourd'hui. Il borne en effet l'interdiction des embryons chimériques l'interdiction des embryons chimériques à la seule modification d'embryons humains avec insertion de cellules provenant d'autres espèces. Ce faisant, il autorise tout ce qui ne correspond pas à cette définition et ouvre donc une nouvelle voie d'expérimentation. Il permet ainsi la création d'embryons chimériques par insertion dans un embryon animal de cellules souches embryonnaires humaines. embryonnaires humaines. La commission spéciale a refusé d'aller plus loin que ce qui est possible aujourd'hui, tout en ajoutant des verrous pour éviter toute dérive. Dans ces conditions, la commission spéciale a réintroduit, à l'article 17, l'interdiction visant l'insertion de cellules souches embryonnaires dans un embryon animal. Pour ce qui est des embryons chimériques recourant aux cellules iPS humaines, outre le respect des principes éthiques fondamentaux, elle encadre leur utilisation à l'article 15, d'une part, en prévoyant l'impossibilité de poursuivre à terme la gestation, et, d'autre part, en fixant une proportion minoritaire de cellules d'origine humaine pour limiter le taux de chimérisme, afin de s'assurer que ces embryons restent bien toujours des embryons animaux. Voilà donc le cadre de notre débat. Ce qui est en jeu, c'est une ligne rouge de la bioéthique à la française, la question du franchissement de la barrière des espèces. Le CCNE a réclamé a réclamé un encadrement de ces expérimentations, car insérer dans un embryon animal ne serait-ce que quelques cellules iPS humaines n'est pas une démarche anodine. C'est à ce besoin d'encadrement que la commission spéciale a cherché à répondre. Ce sera évidemment au Sénat de décider si cet encadrement lui semble pertinent et suffisant. La parole

Cette technique d'édition du génome a récemment bouleversé le monde de la recherche. Elle permet de mettre en oeuvre, au niveau de la cellule, des ciseaux génétiques à base de protéines qui font automatiquement muter des séquences d'ADN, sans injection d'ADN extérieur. Autrement dit, cette technique permet d'introduire un gène à la place d'un autre, ou d'en supprimer. Les ciseaux génétiques créent des mutations facilement et à un coût dérisoire par rapport aux anciennes techniques. Dès lors, on imagine aisément comment leur usage pourrait, à terme, devenir massif dans les laboratoires, même si tous leurs effets biologiques sont loin d'être maîtrisés. Cette technique désormais bien connue révolutionne la fabrication d'OGM. Monsanto en possède une licence d'utilisation pour créer des semences génétiquement modifiées. Fin 2018, en Chine, elle a permis la naissance des premiers « bébés OGM », censément immunisés contre le virus du sida, et cela hors de tout cadre légal, provoquant un scandale planétaire. Le chercheur responsable vient d'ailleurs d'être condamné à trois ans de prison. La levée, même partielle, de l'interdit chimérique et transgénique permettrait à CRISPR-Cas9 de passer officiellement de la semence agricole à l'humain. La nouvelle loi pourrait donc ouvrir la voie à l'industrialisation de la modification génétique des embryons humains à une vitesse encore jamais atteinte. Considérant que cette technique n'a pas de portée médicale potentielle pour soigner des êtres humains déjà nés, on voit mal quelle finalité pourrait découler de cette autorisation de libéraliser la recherche, si ce n'est la possibilité d'engendrer des êtres humains génétiquement modifiés Un tel article mériterait à lui seul un débat philosophique et politique d'ampleur. Le voter à la va-vite dans cette loi ne nous paraît pas raisonnable. Extrêmement mal à l'aise avec les dispositions potentiellement eugéniques de cet article, je plaide donc, avec les membres de mon groupe, pour sa suppression. La

désir des chercheurs de tester les fameux ciseaux CRISPR-Cas9, ou ciseaux moléculaires, pour modifier la descendance génétique.

du Gouvernement sur la question des embryons chimériques et sur la portée de leur interdiction inscrite à l'article 17 du projet de loi. J'ai écouté

la réalité du droit actuel, c'est aussi qu'il ne fixe aucun cadre interdisant de conduire des recherches sur des embryons animaux chimériques.

pour deux raisons. Premièrement, de nombreux mécanismes physiologiques ou pathologiques ne peuvent être compris que par l'utilisation de ce type de techniques,

la question sanitaire est bien évidemment essentielle. Deuxièmement, nous sommes passés d'une époque où le caractère tout génétique prévalait à une époque où nous avons besoin de comprendre plus finement les mécanismes cellulaires fondamentaux, notamment les impacts environnementaux sur ces derniers. Il est important que nous puissions le faire sur des embryons chimériques constitués d'agglomérations de cellules souches

il est totalement interdit, et cela le restera, de créer des embryons à des fins de recherche. De même, il est totalement interdit de réimplanter des embryons qui auraient été manipulés génétiquement, de quelque façon que ce soit.

des recherches qui commencent à être envisagées dans les laboratoires. Aussi, il nous est apparu important que les protocoles de recherche relatifs à ces embryons chimériques

partage l'idée qu'il est inadmissible de créer des embryons à des fins de recherche, tout comme il est inadmissible de réimplanter des embryons génétiquement modifiés, de quelque façon que ce soit. Néanmoins, si nous voulons mieux comprendre

Assassi. Cet amendement de suppression a été excellemment défendu par Guillaume Gontard.

L'objectif de la suppression de cette interdiction est de permettre d'évaluer les effets des techniques d'édition génomique, dont CRISPR-Cas9. L'utilisation de cette technique conduira-t-elle, puisque telle est la question, à des bébés génétiquement modifiés en France ? La réponse est non non ! En effet, le transfert à des fins de gestation des embryons faisant l'objet de recherches est interdit. Cette interdiction figure d'ailleurs à l'alinéa 19 de l'article 14 du projet de loi, que nous aborderons tout à l'heure. Pour ce qui concerne à présent les embryons chimériques, les seules expérimentations aujourd'hui possibles en France sont celles qui consistent à introduire dans un embryon animal quelques cellules iPS humaines.

Cela consiste à désactiver dans l'embryon animal le gène lié à la formation d'un organe particulier et à introduire quelques cellules iPS dans l'embryon animal capable de produire l'organe recherché.

Mme la rapporteure. Madame la ministre, nous avons un point de désaccord. Vous nous laissez entendre que, en l'état actuel du droit, la création d'embryons chimériques à partir de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal est possible, en faisant référence au titre V du livre Ide la deuxième partie du code de la santé publique.

La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. » Il concerne donc bien des chimères à partir de cellules souches embryonnaires qui seraient introduites dans un embryon animal.

aussi rapporteure, et Mme la ministre, c'est la première qui a raison : la loi de 2011, dernière loi bioéthique, dit clairement qu'il est interdit de travailler et de faire des recherches sur les embryons transgéniques et sur les embryons chimériques. C'est écrit en toutes lettres ; si la loi a été modifiée sans que le Parlement le sache, prévenez-nous,

et c'est la version du Gouvernement qui sera réintroduite à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que cela assurera un meilleur encadrement ... Je voudrais surtout dire, à cet instant,

Il n'y a eu aucun eugénisme dans notre pays, que je sache ! On ne nous a pas attendus. Ils ne nous attendent pas. Des comités d'éthique, il y en a partout ; des réflexions, il y en a partout. Nous avons maintenant des corps intermédiaires en la matière, notamment le CCNE et l'Agence de la biomédecine, avec son conseil d'orientation. Ces acteurs intermédiaires, soudain, on ne les écoute plus. On est persuadé qu'ils vont se transformer en savants fous. Un chercheur chinois a inséré un CCR5, un gène qui est censé protéger du VIH, chez un enfant. Il est en prison et mis au ban de la communauté internationale.

qui vise la compétitivité de la France par rapport au reste du monde, ce qui justifierait tous les alignements possibles sur le moins-disant éthique. Je voterai, bien sûr, l'amendement qui a été proposé par le groupe CRCE.

d'abord, il veut laisser penser que sa disposition est conforme à la convention internationale d'Oviedo, qui proscrit justement de modifier la descendance. Eh oui ! Or j'affirme que cette disposition est anti-conventionnelle,

iPS ! Effectivement, le texte de la commission rappelle que l'insertion de cellules pluripotentes iPS

inférieure à 50 %. Si je suis favorable à cette disposition, c'est pour permettre à la recherche d'avancer, tout en l'encadrant. Je le rappelle, actuellement, cette recherche n'est pas interdite. Néanmoins, nous devons prendre des précautions. Est-ce que la simple déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine suffit ? Faut-il un régime d'autorisation ?

et cela m'inquiète. Il est donc bon, parfois, d'inscrire dans la loi un certain nombre d'éléments. Il ne s'agit pas d'une forme de défiance vis-à-vis des chercheurs. J'ai toute confiance dans la recherche. Cependant, j'ai beau avoir confiance dans mes concitoyens, de temps en temps, je leur impose des limites dans la loi.

je n'ai pas voté pour l'ouverture de la PMA aux couples de femmes ou pour l'autoconservation des ovocytes -, je ne voterai pas cet amendement de suppression. Je m'en explique.

vise simplement, au travers de techniques de recherche fondamentale, non pas à déboucher sur la création de nouvelles espèces, mais à permettre le travail sur de nouvelles cellules. Au fond, tout le débat tourne autour des recherches sur les cellules souches embryonnaires, sur les cellules pluripotentes et sur leur implantation au sein d'un embryon animal ; à aucun moment, il ne s'agit de créer des êtres génétiquement modifiés. Je crois qu'il y a confusion entre deux notions qui sont

Cet amendement vise à interdire la création d'embryons chimériques qui pourrait résulter de la modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites.

visant à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques, en imposant deux verrous : d'une part, l'impossibilité de mise à bas et de parturition, ainsi que l'interruption de la gestation dans un délai approuvé par l'Agence de la biomédecine ; d'autre part, la mise en place d'un seuil que la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique ne saurait que la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique ne saurait dépasser. Je veux évidemment rendre hommage à cette volonté de Mme la rapporteure d'instaurer des garde-fous. Mais, au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l'animal d'embryons chimériques hybrides entre l'animal et l'homme soulève toute une série de problèmes et d'interrogations éthiques et morales.

l'article 17, dans sa rédaction présente, dispose bien que la création d'embryons chimériques est interdite, que ce soit dans le cadre de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces, ou de celle d'un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines.

L'histoire retiendra peut-être que le Sénat, aujourd'hui, aura interdit que la recherche conduise à ce que des chimpanzés aient, demain, une intelligence humaine, ou encore à ce que des êtres humains aient des caractéristiques de chimpanzés. Mais ce n'est pas le sujet

Le Conseil d'État, dans son avis sur ce texte, avouait que la révision des lois de bioéthique était un exercice juridiquement semé d'embûches. Nous les avons bien mesurées depuis le début de cet après-midi.

même si j'ai confiance dans le discernement éthique des chercheurs, je considère que le Parlement doit assurer sa mission de contrôle en encadrant ces recherches. J'ai donc déposé plusieurs amendements sur cet article.

En 2016, on a ouvert une dérogation dans la dérogation afin de faciliter la recherche visant à améliorer la PMA. Aujourd'hui, on supprime toutes les conditions. Quelle est la prochaine étape ?

N'est-ce pas le constat d'un échec ? Quel est le bilan de ces recherches ? Pourquoi ne pas privilégier les cellules pluripotentes induites, qui sont, selon l'Académie nationale de médecine, l'Agence de la biomédecine et l'Inserm, tout aussi efficaces que les cellules souches embryonnaires humaines ?

qu'une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon humain en soi, le législateur ne peut oublier qu'elle en émane et que son prélèvement en provoque la destruction. article soulève de nombreuses questions, qui sont d'ordre non pas scientifique, mais sociétal. La France veut-elle produire des enfants génétiquement modifiés ? La levée de l'interdit de créer des embryons transgéniques permettra la création en laboratoire d'embryons humains génétiquement modifiés. La responsabilité des politiques est grande, d'autant qu'il n'y a eu aucun débat digne de ce nom sur la fécondation à trois parents ou le ciseau moléculaire. Le Gouvernement essaie de nous rassurer en posant un interdit sur le transfert à des fins de gestation d'embryons génétiquement modifiés, mais l'expérimentation en laboratoire a-t-elle une autre finalité que d'aboutir, à terme, à une expérimentation clinique ?

Ce projet de loi déploie un arsenal juridique considérable pour favoriser la recherche afin de lutter contre l'infertilité. Ce problème, de plus en plus prégnant dans nos sociétés modernes, concerne près d'un couple sur huit dans notre pays. dès lors dommageable que rien, ou presque, dans ce texte n'ait trait à la recherche sur les causes de l'infertilité ou de certaines malformations foetales. Les députés se sont timidement emparés du sujet, mais l'on reste loin du compte Pourtant, si les causes environnementales de l'infertilité sont identifiées, elles ne sont pas parfaitement comprises. Je pense tout particulièrement aux perturbateurs endocriniens, aux ondes électromagnétiques et aux pesticides, toutes choses dont on connaît ou suspecte les effets fertilité du sperme, endométriose, bébés sans bras, et j'en passe ! Ainsi, selon les données de l'Inserm, pour 25 % des couples qui consultent, la science n'est pas en mesure de déceler les causes de l'infertilité. Un couple sur quatre qui ne peut pas avoir d'enfant ne saura pas pourquoi Alors que nous dépensons un temps et un argent considérable à la recherche visant à soigner ou à pallier l'infertilité, il faudrait orienter une partie de cet effort vers la recherche sur ses causes. Un esprit méfiant verrait une explication simple à ce choix unidimensionnel du Gouvernement : prévenir les problèmes de santé est bien moins lucratif pour les laboratoires pharmaceutiques que les soigner. Pour ma part, j'y vois une nouvelle preuve de l'incapacité de l'humanité à accepter les conséquences délétères de son mode de vie sur notre environnement et sur notre propre santé. Comme pour le réchauffement climatique, nous préférons fuir en avant : on dépense une énergie considérable à chercher des palliatifs, plutôt que d'agir pour tenter de corriger les problèmes à la source. Ainsi, de la même manière que l'on invente des bateaux pour nettoyer le plastique des océans ou que l'on cherche un moyen de stocker le carbone, on tente de corriger, à grand renfort de manipulations génétiques, les causes de l'infertilité, alors qu'il conviendrait en premier lieu de cesser de produire du plastique jetable, de diminuer les émissions de carbone et de se débarrasser des perturbateurs endocriniens et autres pesticides. C'est pourquoi nous défendrons un amendement relatif, notamment, à la recherche sur les perturbateurs endocriniens. Je

aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires. Compte tenu des enjeux de ce type de recherche et, notamment, de l'industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l'Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en oeuvre.

voire l'industrialisation de la production de ces cellules souches embryonnaires est l'un des enjeux du business de l'industrie pharmaceutique. Rendre ainsi disponibles ces cellules peut susciter un risque majeur d'industrialisation de de l'humain. Au regard de l'atteinte portée à l'embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, il est nécessaire que l'Agence de la biomédecine, garante du cadre légal et des principes éthiques, mène en amont une instruction sur les protocoles de recherche. En somme, nous proposons au travers de cet

que pour instituer un délai limite de culture des embryons surnuméraires, délai qui n'existe pas aujourd'hui. Par ailleurs, cette suppression reviendrait sur la mise en place d'un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place de l'actuel régime d'autorisation. Or si le projet de loi procède à une différenciation des régimes juridiques applicables aux recherches sur l'embryon et à celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires, c'est précisément pour acter la différence de nature entre l'embryon et les cellules souches qui en sont issues. Une fois dérivées d'un embryon, les cellules souches n'ont pas la capacité d'en former spontanément un nouveau. Elles n'ont en rien le caractère symbolique de la personne potentielle qu'on attribue à l'embryon, comme l'a rappelé le Comité consultatif national d'éthique. De plus, une fois qu'elles sont constituées, les lignées de cellules souches embryonnaires n'impliquent plus la destruction d'un embryon. Dans ces conditions, le maintien d'un régime d'autorisation analogue à celui qui est applicable aux recherches sur l'embryon ne se justifie plus, éthiquement, pour les recherches qui portent sur les cellules souches embryonnaires.

surtout quand il s'agit de recherche sur les embryons. On compte actuellement 19 000 embryons, dont, en l'absence de projet parental, on a proposé

les deux pieds sur terre ! Leur vocation est bien d'aller trouver une innovation médicale qui soit acceptable par

pense aux recherches sur l'infarctus du myocarde et sur certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou la chorée de Huntington -trouvent potentiellement leur origine dans cette phase embryonnaire.

Ces déclarations ont poussé le Parlement à consentir des dérogations, puis à autoriser les recherches sur l'embryon et les cellules souches. En 2011, on nous disait que les cellules souches embryonnaires humaines permettraient de créer des pansements provisoires pour les grands brûlés. En 2013, on nous disait que l'on était sur le point de guérir les patients

nécessitent-elles des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ? Il n'y a aucune thérapie effective en la matière. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quel bilan peut-on dresser de ces dérogations et autorisations ?

les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines dans l'attente d'une évaluation de ces recherches par l'Opecst. Or la loi charge déjà l'Agence de la biomédecine d'évaluer, dans son rapport annuel d'activité, l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, en incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu'un comparatif avec la recherche internationale.

entre le moment où l'on entame des recherches et celui où l'on aboutit à un médicament, il y a évidemment, et fort heureusement, un certain nombre d'étapes, qui sont essentielles

ou le traitement des maladies métaboliques du foie. Je mentionnerai également deux projets, qui ont permis d'identifier des molécules utilisées dans des essais cliniques sur des patients atteints d'une forme génétique d'autisme et de la myotonie de Steinert, qui est une maladie génétique orpheline. deux projets qui visent à élucider les mécanismes permettant de comprendre la pluripotence et à découvrir si, de la même façon que nous avons maintenant des cellules souches pluripotentes induites, nous pourrions avoir d'autres

J'ai un léger souci avec la rédaction de l'alinéa 2, qui dispose que les recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation « peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu avant ou

on lit exactement le contraire : « Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite, en application du présent article, ne peuvent être transférés à des fins de gestation. » Cela n'a rien à voir ! Mon amendement a pour objet de tenter de mettre en cohérence l'alinéa 2 avec l'alinéa 19

aux recherches interventionnelles. Seules les recherches observationnelles dénuées de risques sont envisageables et éviteront la manipulation génétique des gamètes ou des embryons. Tel est le sens de cet amendement de précision. L'amendement n° 187, présenté par M.

l'article 16-4 du code civil, « nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine », et l'article 16-2 du même code rappelle que « le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher [ ...] les agissements illicites portant sur des éléments ou des produits » du corps humain. Or les gamètes sont des cellules particulières, obtenues après un long processus dans les gonades, favorisant la réalisation, à partir de cellules précurseurs, du phénomène de méiose, qui permet un brassage génétique favorable à l'espèce humaine, ainsi que le passage de quarante-six à vingt-trois chromosomes. Il convient donc de rappeler l'interdiction d'un processus intégrant une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.

procréation médicalement assistée sont autorisées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), seulement pour celles qui ont un caractère interventionnel à risque. Ces autorisations ne sont pas publiées au. Il s'agit Il s'agit aujourd'hui de recherches dont on ne sait rien : on ne connaît ni la nature des travaux qui ont pu être menés depuis trois ans, ni leur finalité, ni, enfin, le résultat obtenu. La manipulation des gènes peut constituer un vrai danger, dans la mesure où les modifications génétiques peuvent avoir des répercussions sur plusieurs générations.

il me semble plus que légitime de mettre en place une mission d'information, qui permettra de faire le bilan des travaux menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans, et de savoir s'ils ont été implantés. Après tout, c'est la mission du Parlement que d'assurer ce contrôle.

conduites « en application du présent article ».

De fait, tout risque pour l'embryon ne peut, dans l'absolu, être écarté dans le cadre d'un essai clinique, comme c'est le cas pour tout autre essai clinique interventionnel, notamment lorsque l'essai consiste à expérimenter un milieu de préparation de cultures destinées à favoriser la maturation et l'implantation de l'embryon. Dans ce cas, la recherche sera assortie de toutes les garanties qui s'attachent aux recherches biomédicales et ne sera entreprise qu'avec l'autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Celle-ci se prononcera notamment au regard du caractère satisfaisant

les recherches menées sur l'embryon dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation sont nécessairement considérées comme des recherches interventionnelles, et ce pour deux raisons. elles impliquent un transfert dans l'utérus de la femme et comportent, donc, à tout le moins, une intervention sur cette dernière. Par ailleurs, plusieurs recherches autorisées dans ce cadre par l'ANSM ont pu impliquer des interventions sur l'embryon par l'expérimentation de milieux de culture favorisant une meilleure maturation ou une meilleure implantation,

défavorable. L'amendement n° 187 tend à inscrire l'interdiction de la différenciation de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites en gamètes dans les dispositions relatives aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Or ces recherches ne peuvent en aucun cas donner lieu à ce type d'expérimentation : elles portent uniquement sur des gamètes issus de donneurs tiers ou du couple candidat à l'AMP, ou sur l'embryon constitué dans ce cadre.

pour dresser le bilan des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Une audition de l'ANSM sur l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat serait probablement un meilleur moyen de mettre un coup de projecteur sur un tel bilan. Au reste, les résultats des essais cliniques autorisés par l'ANSM et conduits dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation sont ou seront disponibles en fonction de l'état d'avancement de la recherche sur le site clinicaltrials.gov. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission spéciale demande à son auteur de bien

Tout d'abord, il ne faut absolument pas confondre la recherche menée sur des embryons, pour lesquels il n'y a plus de projet parental et qui ont vocation à être détruits, la recherche menée dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, qui est un acte médical ayant pour objet de favoriser la grossesse. Cette distinction est très claire dans la loi, et ces dispositions ne figurent pas du tout

n'impliquant pas de modèles animaux, car ils nous permettront de mieux comprendre la différenciation des gamètes et, donc, potentiellement, de trouver des solutions aux problèmes d'infertilité. Le Gouvernement

rectifié , la loi en vigueur rend effectivement possibles les recherches interventionnelles et observationnelles sur l'embryon. Mon amendement vise justement à ne permettre que les recherches observationnelles, qui sont dénuées de risques, donc à interdire les recherches interventionnelles qui, elles, sont à risque.

Les recherches conduites dans le cadre de la prise en charge médicale de personnes ayant recours à une assistance médicale à la procréation sont des essais cliniques et relèvent du régime des recherches impliquant la personne.

humaine. L'article L. 1125-3 du code de la santé publique modifié figure dans un chapitre intitulé « Dispositions particulières à certaines recherches », au sein du titre spécifiquement consacré

Depuis 2016, c'est le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui est chargé d'autoriser les recherches biomédicales en PMA. Ces recherches, qui portent sur l'embryon humain, ne sont pas publiées au. C'est C'est d'autant plus étonnant que les autorisations de recherche sur l'embryon qui sont, elles, délivrées par l'Agence de la biomédecine, sont publiées au. Je vous rappelle que les recherches biomédicales menées dans le cadre d'une PMA portent sur l'embryon humain, au même titre que celles qui sont menées dans le cadre de la recherche

spéciale ? Tous les protocoles de recherche autorisés par l'ANSM, dont ceux qui portent sur l'embryon dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, sont déjà publiés sur le site de référence clinicaltrials.gov, qui est d'accès libre. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre des règlements européens relatifs aux essais cliniques, un portail européen sera bientôt mis en place pour regrouper toutes les informations et données relatives aux essais autorisés. Pour ces raisons, l'avis de

sur les cellules souches embryonnaires. Son adoption conduirait, en réalité, à restaurer un régime d'autorisation préalable par l'Agence de la biomédecine pour la mise en oeuvre des recherches sur ces mêmes cellules. Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l'embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires, qui ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques. En effet, une fois dérivées, les cellules souches embryonnaires n'impliquent plus la destruction de l'embryon et ne sont pas en capacité de former spontanément un nouvel embryon, comme nous l'observions précédemment. Un régime de déclaration préalable pour ces recherches, avec un pouvoir d'opposition que l'Agence de la biomédecine peut exercer dans un délai fixé par voie réglementaire, si elle constate la méconnaissance de certains prérequis et des principes éthiques fondamentaux, apparaît donc plus pertinent. L'avis de la commission spéciale est donc défavorable.

spéciale ? Au considérant 10 de sa décision relative à la loi de 2013 ayant modifié le régime juridique des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, le Conseil constitutionnel a rappelé que les principes éthiques applicables à ces recherches découlent des « principes fixés notamment aux articles aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés, et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain Les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires humaines sur lesquels des recherches peuvent être pratiquées doivent en effet avoir été produits dans un cadre respectueux de la dignité du corps humain, encadré, justement, par les articles 16 à 16-8 du code civil. Ces articles impliquent non seulement l'interdiction des pratiques eugéniques et du clonage, figurant à l'article 16-4, mais également l'inviolabilité du corps humain- article 16-1 -, le consentement de la personne à toute intervention sur son corps et les éléments qui en sont issus- article 16-3 -et l'impossibilité pour ces éléments de faire l'objet d'un droit

Legge. Le projet de loi tend à supprimer l'évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur, ainsi que de l'information qui lui revient. Autrement dit, on supprime l'obligation faite à l'Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur

? L'adoption de cet amendement conduirait à mettre en place une information systématique du couple ayant cédé ses embryons à la recherche sur la nature des recherches susceptibles d'y avoir recours. Or l'article R. 2151-4 du code de la santé publique prévoit déjà qu'« une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5 est délivrée ».

Un document d'information et de consentement leur est transmis, indiquant les choix qui leur sont ouverts, et l'Agence de la biomédecine édite un modèle de documents à cet effet.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, une nouvelle disposition a été adoptée, permettant aux membres d'un couple de se prononcer de manière anticipée sur la possibilité

La limite de quatorze jours correspond à un événement majeur du développement embryonnaire : la gastrulation. Cet événement aboutit à la mise en place des trois feuillets embryonnaires qui seront à l'origine de l'ensemble des organes l'ectoderme, à l'origine de la peau et du système nerveux ; le mésoderme, qui formera les muscles ou le squelette ; l'endoderme, à l'origine du tube digestif ou des voies respiratoires. La séparation de ces trois feuillets aboutit à la formation de la ligne primitive, qui donnera plus tard, au dix-neuvième jour, l'ébauche du tube neural et des futures cellules nerveuses. La limite de quatorze jours est donc regardée comme marquant l'apparition des premières ébauches du système nerveux central.

n° 248 rectifié . Le développement d'embryons à des fins de recherche doit être soumis au critère du développement des premières cellules nerveuses chez l'embryon. Or, le consensus scientifique s'établit sur une limite de quatorze jours. Il n'est donc pas souhaitable

dans un rapport qui fait encore référence de nos jours. Elle a été retenue par de nombreux autres États. Comme cela a été particulièrement bien expliqué, elle correspond au stade où apparaissent les premières ébauches du système nerveux et où l'embryon s'individualise réellement : c'est effectivement à partir de ce stade qu'il ne peut plus se scinder pour donner de vrais jumeaux. Il ne nous semble donc pas souhaitable d'aller au-delà de cette limite de quatorze jours, celle-ci ouvrant déjà la voie à un approfondissement

! Une meilleure compréhension des étapes du développement embryonnaire entre le quatorzième et le vingt et unième jour, qui concernent effectivement la période dite de gastrulation, présente un intérêt scientifique majeur. Les scientifiques insistent sur l'importance d'étudier ces mécanismes de développement chez l'embryon humain, afin de mieux appréhender le contrôle de la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines et pluripotentes induites, ainsi que les retombées médicales potentiellement associées. Ces mêmes scientifiques ont mis en avant le fait que cette troisième semaine, c'est-à-dire la phase de gastrulation, est une période critique, au cours de laquelle environ 20 % des grossesses s'arrêtent spontanément à la suite d'une anomalie du développement embryonnaire. Comprendre les causes de ces anomalies du développement embryonnaire et apprendre à les prévenir constitue donc un enjeu important. D'où la nécessité, pour la commission spéciale, de permettre aux scientifiques de se pencher sur le sujet.

Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d'un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient d'appliquer le même régime commun de sept jours pour la durée de conservation.

les prérequis demandés pour la recherche sur l'embryon ne s'appliqueraient plus à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Il ne serait plus nécessaire que la pertinence scientifique de la recherche soit établie. La recherche,

à M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement tend à cantonner le régime de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux lignées déjà existantes. Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l'embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes.

La recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l'étranger. Cela permet de résoudre le conflit éthique associé à la dérivation de nouvelles lignées, qui implique la destruction d'embryons humains. Les lignées de cellules souches embryonnaires humaines sur lesquelles les chercheurs travaillent dans le monde et en France sont connues. Elles peuvent donc faire l'objet d'une liste, qui permettra de limiter ces recherches aux seules lignées déjà existantes. Quel est l'avis spéciale ? S'agissant de l'amendement n° 178, l'agrégation de cellules souches embryonnaires à des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires conduit à la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes. Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer certaines fonctionnalités embryonnaires, ils feront précisément l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'Agence de la biomédecine : celle-ci pourra en effet s'opposer à tout protocole de ce type qui violerait les principes éthiques fondamentaux, avec, systématiquement, un avis public de son conseil d'orientation.

autorisé par l'Agence de la biomédecine ou d'avoir été importées dans le cadre d'une autorisation d'importation également délivrée par l'Agence de la biomédecine. Or ces autorisations permettent précisément de garantir que les cellules souches embryonnaires utilisées ont été dérivées dans des conditions respectueuses de nos principes éthiques. Supprimer cette obligation reviendrait à permettre des recherches à partir de cellules souches embryonnaires ne présentant pas ces garanties éthiques. La commission spéciale demande donc viens à l'amendement n° 78 rectifié . Le fait de limiter les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées déjà existantes aurait pour effet de restreindre considérablement les potentialités de telles recherches. En effet, cela conduirait à exclure la possibilité de mener des recherches sur des lignées de cellules souches embryonnaires nouvellement dérivées, à partir d'embryons présentant des caractéristiques jusqu'ici inconnues, comme, par exemple, une anomalie génétique tout juste identifiée. Pour ces raisons, de nouveau, l'avis de

de l'amendement n° 79 rectifié , toutes les lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles en Europe, donc en France, sont répertoriées dans le registre européen des cellules souches pluripotentes humaines, accessible à tous. Il n'y a donc pas lieu d'acter par décret l'existence de ces lignées. La commission spéciale

les recherches autorisées par l'Agence de la biomédecine sont réalisées sur des cellules souches embryonnaires humaines dérivées voilà plusieurs années. Ainsi, Mme Cécile Martinat, chercheur sur les cellules souches embryonnaires et présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches, soutenait lors de son audition devant notre commission spéciale : « Cela fait bien longtemps que l'on n'a pas dérivé de cellules souches embryonnaires humaines. Cela fait un peu plus de 15 ans que je travaille sur ces cellules. Je n'ai jamais détruit un embryon. J'utilise des lignées qui ont été dérivées voilà maintenant 20 ans. L'Allemagne, elle, cantonne sa recherche sur l'embryon aux lignées de cellules souches embryonnaires humaines importées ; elle n'est pas pour autant en retard dans ce domaine de recherche. » Il semble donc opportun de faire de la recherche exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes. Je maintiendrai donc cet amendement.

L'utérus artificiel est d'ailleurs aujourd'hui techniquement possible et, à l'étranger, son expérimentation est en cours. C'est notamment le cas aux États-Unis, en Angleterre et en Israël, où des chercheurs ont déjà réussi à modéliser une paroi utérine humaine. Le fait, en parallèle, que la France repousse la limite de conservation des embryons humains jusqu'à vingt et un jours ne peut que rendre plus utile l'interdit de l'utérus artificiel, pour éviter toute tentation de conserver plus longtemps l'embryon humain. cette technique en France, « sans doute cette technique aura-t-elle d'abord des fonctions thérapeutiques, remplaçant les incubateurs actuels pour maintenir en vie les grands prématurés. Mais personne n'est dupe. [ ...] Comme les inséminations artificielles et les fécondations, les utérus artificiels seront utilisés pour des " désirs d'enfant " que la procréation naturelle, non médicalisée, ne permet pas de satisfaire.

l'avis de la commission spéciale ? Cette interdiction de l'expérimentation de l'utérus artificiel ne me paraît pas appropriée à cet endroit du texte, car l'alinéa 19 prévoit déjà explicitement que les embryons surnuméraires ayant fait l'objet d'une recherche ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Ils ne pourront donc pas,, être transférés dans un utérus artificiel. Par ailleurs, je rappelle que, lorsque des recherches sont menées sur un embryon dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, elles relèvent des recherches biomédicales et ont pour objectif un transfert de l'embryon chez la femme. Ces embryons ne peuvent donc pas faire l'objet d'un transfert dans un utérus artificiel. Lorsque des recherches sont menées sur des embryons surnuméraires, le transfert à des fins de gestation est, lui, interdit.

Nous le déplorons, et souhaitons, sinon ouvrir la possibilité pour la recherche de se pencher sur ce sujet, du moins l'encourager, notamment en ce qui concerne les conséquences des perturbateurs endocriniens et des ondes électromagnétiques sur l'infertilité. En effet, ne serait-il pas plus logique de réfléchir à l'infertilité en la traitant par ses causes et non par ses conséquences ? Or rien n'est fait en ce sens, aucune recherche n'est réalisée sur les facteurs environnementaux- pesticides, pollution, perturbateurs endocriniens -ou sur le mode de vie- tabagisme, sédentarité, etc.

À ce jour, sur les 23 protocoles de recherche sur l'embryon qui ont été autorisés par l'Agence de la biomédecine, 9 concernent l'étude du développement embryonnaire préimplantatoire, avec un lien direct sur sa qualité ou la capacité d'implantation de l'embryon. Par ailleurs, l'Agence de la biomédecine autorise les protocoles de recherche sur la base de critères objectifs, notamment au regard de leur pertinence scientifique ; en revanche, elle n'a pas vocation à les hiérarchiser selon leur objet. Elle n'a, de toute façon, aucun moyen d'encourager un type de recherche par rapport à un autre.

par cette proposition, vous souhaitez appeler l'attention sur la nécessité de mener des recherches sur les causes de l'infertilité, ce qui ne peut qu'être approuvé.

rectifié. En parallèle à nos débats, qui ont porté tant sur l'extension de la PMA que, à l'instant, sur les recherches sur l'embryon, il me paraît nécessaire de considérer plus en détail les raisons qui amènent à constater une hausse des situations infertilité.

Les familles concernées souhaitent que la puissance sanitaire publique approfondisse ses investigations en s'intéressant à l'effet cocktail ou multifactoriel, par exemple. Dans ce flou,

désemparés. Nous devons être attentifs aux attentes de la population. Il est du devoir de l'autorité sanitaire publique d'y répondre, faute de quoi la tentation sera grande, pour les proches des malades ou les parents des bébés, de confier à des laboratoires privés

des études alarmantes ont conclu, notamment en Occitanie et plus particulièrement à Toulouse, que la qualité des spermatozoïdes a été divisée par trois chez les hommes trentenaires. Il faut regarder le problème en face et ne pas se

Dès lors qu'un embryon humain porteur même d'une seule cellule animale est interdit- c'est une bonne chose -, il est important de contrôler que l'adjonction de cellules humaines dans un embryon animal, par le biais des procédures autorisées par l'article 17, qui a maintenant disparu, ne conduise pas à des organismes, même embryonnaires ou foetaux, dont le statut d'espèce serait indéfini. Le Comité consultatif national d'éthique d'éthique précise en outre, dans son avis 129, que de telles expérimentations pourraient « faire l'objet d'une évaluation et d'un encadrement par une instance [ ...], si ces embryons sont transférés dans l'utérus d'un animal Dans cet esprit, le présent amendement a pour objet de soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations, dès lors qu'un transfert chez la femelle d'un embryon chimérique est envisagé, en mettant en place un régime propre d'autorisation, subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la commission spéciale au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d'autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l'embryon humain. Dans la mesure où l'Agence de la biomédecine sera chargée de définir les délais de gestation autorisée et les seuils des pourcentages de cellules humaines dans l'embryon chimérique

et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d'autorisation par l'Agence de la biomédecine. C'est au regard des garanties effectives apportées par ces autorisations que le Conseil constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision du 1 août 2013, que les dispositions de ce régime « ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne ». Or l'article 14 dissocie les régimes applicables respectivement à la recherche sur l'embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines. En substituant un régime de déclaration à un régime d'autorisation, cet article crée un régime de recherche, sur les cellules souches embryonnaires humaines, qui soit distinct du régime de recherche sur l'embryon humain. sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l'embryon pour ne les soumettre qu'à une simple déclaration est une proposition qui ne tient pas compte de la réalité ontologique de l'embryon humain. Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle, en les livrant à l'industrialisation. Au regard de l'atteinte portée à l'embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, il apparaît nécessaire que l'Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en oeuvre. Le présent amendement tend donc à maintenir le régime commun, qui repose sur une autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine, tel qu'il est actuellement applicable aux deux types de recherche, sur l'embryon, d'une part, et sur les cellules souches embryonnaires humaines, d'autre part.

le rétablissement d'un régime d'autorisation préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place du régime de déclaration prévu par le projet de loi. de l'amendement n° 151 rectifié, la suppression de l'article 17 revient à supprimer la création d'embryons chimériques, soit par l'introduction de cellules souches embryonnaires humaines

Concernant les amendements identiques n 56 rectifié et 131 rectifié , la mise en place d'un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires permet effectivement d'acter la différence de nature entre ces dernières et l'embryon. J'ai eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois, une fois dérivées, les lignées de cellules souches embryonnaires ne sont pas capables de constituer spontanément un embryon. Les recherches portant sur ces cellules ne soulèvent donc pas les mêmes enjeux éthiques que l'intervention sur l'embryon. Le régime d'autorisation des recherches sur l'embryon se justifie en grande partie par le fait qu'elles impliquent à un moment sa destruction. Toute dérivation d'une lignée de cellules souches embryonnaires, bien qu'elle implique la destruction de l'embryon, reste cependant bien soumise, cela a aussi été dit précédemment, à un régime d'autorisation, puisqu'il s'agit d'une opération conduite sur un embryon.

spéciale ? Le maintien du prérequis de l'absence de méthodologie alternative n'est pertinent que pour les recherches sur l'embryon, et non pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. En effet, celles-ci ne présentent plus les mêmes propriétés qu'un embryon, puisqu'elles n'ont pas la capacité de former spontanément un nouvel embryon. En outre, ce prérequis a eu jusqu'ici pour effet de fragiliser les protocoles de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines, puisqu'il laissait entendre que le recours aux cellules pluripotentes induites pouvait constituer une solution de rechange pertinente. Or l'on sait désormais que, si elles sont proches,

L'Agence se voit ainsi privée de son pouvoir de décision et de contrôle, qui est si important au vu des enjeux. Cet amendement vise donc à le rétablir. Quel est l'avis de la commission Outre que ses dispositions présentent une incohérence, cet amendement vise à soumettre des recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires à une procédure d'autorisation préalable. Pour ce faire, il tend à renvoyer au régime d'autorisation applicable aux recherches sur l'embryon. Or les recherches sur l'embryon et celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires font l'objet de régimes distincts, inscrits désormais par le projet de loi à deux articles différents du code de la santé publique. Il ne suffit donc pas de faire référence au régime applicable à l'embryon pour le rendre applicable aux cellules souches embryonnaires.

L'Agence peut en effet s'opposer à ces protocoles si elle estime qu'ils violent les principes éthiques fondamentaux, et, dans ce cas, la décision d'opposition sera systématiquement précédée d'un avis public de son conseil d'orientation. Je rappelle que la recherche sur les cellules souches embryonnaires n'est possible à partir d'embryons

L'amendement n° 135 rectifié vise à préciser que les gamètes obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une fécondation pour constituer un embryon. La commission spéciale a d'ores et déjà précisé que la création d'embryons par fusion de gamètes, quelle que soit l'origine de ces derniers, est interdite. Bien qu'elle soit redondante, la précision apportée par l'amendement peut néanmoins permettre d'insister sur l'interdiction absolue de constituer des embryons à des fins de recherche. C'est la raison

2004. Elle figure donc déjà parmi les grands principes éthiques qui guident nos réflexions et n'a pas été modifiée. Cela s'applique bien évidemment aux recherches sur les cellules souches embryonnaires comme aux recherches sur les cellules souches pluripotentes induites. Votre demande est donc satisfaite,

à M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement tend à prévoir que l'importation de cellules souches embryonnaires humaines ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d'Oviedo. Il est en effet étonnant que de nombreuses autorisations d'importation délivrées par l'Agence de la biomédecine portent sur des lignées de cellules souches provenant des États-Unis, d'Israël, d'Angleterre, autant de pays qui ont refusé de signer la convention d'Oviedo, dont l'article 18 a pour objet, je le rappelle, de protéger Ces pays sont dotés d'une législation moins protectrice de l'embryon que la France. Pour éviter un contournement de la loi française ou internationale qui constituerait une fraude à la loi, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu'elle, et non de pays moins-disants éthiques.

le code de la santé publique prévoit déjà que l'importation de ces cellules souches ne peut être autorisée par l'Agence de la biomédecine que si elles ont été obtenues dans le respect des principes éthiques fondamentaux prévus par notre législation, principes qui découlent précisément de la convention d'Oviedo. Que des lignées soient importées de pays n'ayant pas signé ou ratifié la convention d'Oviedo n'implique pas en effet nécessairement que ces lignées aient été produites en méconnaissance des principes éthiques posés par cette convention. Chaque fois qu'elle autorise une importation de cellules souches embryonnaires, l'Agence de la biomédecine vérifie que ces cellules ont bien été obtenues dans le respect des principes éthiques. À titre d'information, dans son rapport d'activité publié en 2019 et concernant l'année 2018,

C'est ce que nous réaffirmons dans le projet de loi, et tel est l'objet du contrôle rigoureux exercé par l'Agence de la biomédecine avant toute autorisation d'importation. En restreignant le droit d'importer des lignées de cellules souches embryonnaires aux seuls États signataires de la convention d'Oviedo, priverait les équipes de recherche françaises de la possibilité d'utiliser des lignées qui font référence partout dans le monde et qui- le fait est attesté -respectent les exigences éthiques. J'émets donc un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

pour le projet de loi organique relatif au système universel de retraite et pour le projet de loi instituant un système universel de retraite. Tiens donc ! C'est un scoop

prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 22 voix pour, 3 voix contre et 5 bulletins blancs -à la nomination de M. Didier Migaud aux fonctions de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.